Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

au cours duquel Yann, Alain et Dimitri, trois sauveteurs en mer, ont perdu la vie lors d'une opération de sauvetage d'un bateau de pêche. Ce drame a été à l'origine de la création de la mission commune d'information sur le sauvetage en mer et la sécurité maritime. C'est une décision de la conférence des présidents, prise sur l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, qui a permis la constitution de cette mission très rapidement, dès le 9 juillet 2019. L'événement tragique du mois de juin avait provoqué une émotion immédiate de l'opinion publique et des hommages sincères de la part de tous les responsables locaux et nationaux. Notre mission avait pour objet d'aller plus loin, de dépasser la réaction compassionnelle pour comprendre comment cet accident, où l'état du matériel a tenu une part déterminante,

En parfait accord avec Corinne Féret, présidente de la mission- je la remercie du soutien qu'elle m'a apporté et de la très bonne ambiance qui a régné tout au long de nos travaux -, la mission d'information a décidé de travailler selon une méthode assez particulière. Tout d'abord, nous avons privilégié l'écoute des intervenants du terrain au format plus convenu des auditions au Sénat. Ainsi, le programme de nos déplacements- douze au total -a conduit des délégations de sénateurs à se rendre en Vendée- aux Sables-d'Olonne, où un hommage a été rendu aux sauveteurs disparus -, puis dans les départements des Alpes-Maritimes, du Calvados, de la Manche, du Finistère, de Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, ainsi qu'en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. À ce titre, je remercie Jean-François Rapin et Michel Vaspart qui, à la faveur d'un déplacement, ont représenté notre mission en ces contrées lointaines. À chaque fois, nous avons recueilli les témoignages et les remarques de l'ensemble des intervenants bénévoles de la SNSM, canotiers, patrons, présidents et trésoriers des stations, responsables des centres de formation et du pôle de soutien technique de la flotte, délégués départementaux, inspecteurs, élus locaux, responsables des centres régionaux Ce n'est qu'à l'issue de ces rencontres, qui nous ont beaucoup appris, que nous avons réalisé les auditions des responsables institutionnels en clôturant par le témoignage de deux des rescapés du drame du 7 juin La seconde particularité a été la célérité. Les missions d'information disposent traditionnellement de six mois pour présenter leurs conclusions. Nous avons mené nos travaux en trois mois et demi, en utilisant au maximum la période estivale pour nos visites dans les stations et les centres de formation.

Au terme de ses travaux, la mission d'information a établi une liste de trente propositions réparties en trois grands axes : mieux reconnaître le bénévolat et son engagement humaniste, garantir sur le long terme le financement des investissements et, enfin, démocratiser le fonctionnement de la SNSM et clarifier la répartition des rôles. Ces propositions résultent bien sûr de notre réflexion. Mais elles reprennent aussi des demandes, parfois très modestes, qui nous ont été faites lors de nos déplacements et qui ont une forte valeur, une forte portée symboliques. Sur chacun des trois thèmes, je reprendrai les propositions qui me paraissent les plus importantes. La mission d'information n'a jamais remis en question le principe du bénévolat, qui est en réalité l'ADN du sauvetage en mer. Mais les sauveteurs bénévoles ressentent un manque de reconnaissance de la Nation, auquel il convient de répondre par des mesures concrètes. Avant tout, la mission appelle donc à un travail avec les employeurs des sauveteurs. Ce travail devrait viser, d'une part, à améliorer le cadre de la disponibilité des sauveteurs pour leurs interventions et, d'autre part, à renforcer l'accès des sauveteurs à la formation, le droit individuel à la formation Aujourd'hui les bénévoles sont trop souvent laissés seuls pour négocier directement avec leurs employeurs. À nos yeux, c'est au délégué départemental de la SNSM de recenser leurs demandes et de faire la démarche auprès des employeurs des sauveteurs pour formaliser des conventions leur permettant d'être plus facilement détachés de leurs obligations professionnelles dès lors qu'ils sont appelés à intervenir Ce sont bien toutes les institutions qui doivent mieux reconnaître le bénévolat, l'État comme les organismes de formation et, bien sûr, la SNSM. La mission préconise ainsi l'accès aux congés de formation, l'octroi de jours de délégation pour certains cadres de la SNSM, la reconnaissance d'équivalence et l'uniformisation des diplômes de formation entre le ministère de l'intérieur, le ministère de la santé et la marine marchande. marchande. En outre, la mission considère que tous les bénévoles devraient être adhérents de la SNSM, alors qu'aujourd'hui ils n'ont aucun rôle reconnu dans la gestion de cette association. Au titre du financement, deux points me paraissent essentiels.

en réduisant autant que possible leurs frais de fonctionnement. Ainsi, le gros entretien des navires absorbe souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors même que les stations peinent à s'alimenter en carburant pour assurer les sorties en mer.

D'une part, l'affectation à la SNSM de taxes existantes, comme la fiscalité des permis de plaisance ou le produit des redevances de l'État sur l'occupation du domaine public maritime. D'autre part, le déploiement d'incitations fortes pour que l'ensemble des usagers de la mer, de plus en plus nombreux et divers, participent au financement du sauvetage en mer. Nous avons envisagé, en ce sens, la création d'une contribution volontaire à l'achat de navires neufs et d'engins et matériels nautiques- paddles, kitesurfs, kayaks de mer, planches à voile, etc. -, dont le montant serait progressif en fonction du coût de l'équipement. Enfin, pour ce qui concerne la gouvernance, les recommandations de la mission sont parties d'un constat : les bénévoles des stations et le siège de la SNSM sont aujourd'hui deux mondes qui ne se comprennent et ne se parlent plus. Cette situation est due en grande partie au caractère pyramidal, centralisé et peu démocratique de la SNSM, institution, et même « vache sacrée », selon les termes mêmes de son ancien président, qui peine à se réformer. Nous en sommes convaincus : la SNSM aurait tout intérêt à s'inspirer de l'organisation de la protection civile. Ce serait là un moyen de rendre plus attractif le recrutement des bénévoles, enfin considérés comme de véritables acteurs de leur association. Cette évolution implique de reconnaître dans les statuts de la SNSM la notion d'adhérent dans la plénitude de ses attributions. Elle devrait conduire, dans l'idéal, à adopter une structure fédérale- la SNSM deviendrait ainsi une fédération regroupant des associations départementales affiliées.

Le bilan a été fait de notre système de sauvetage. Le rapport de la mission d'information n'est d'ailleurs pas le premier à l'avoir établi. En effet, deux rapports précédents le relevaient déjà : notre système obtient d'excellents résultats pour un coût minime pour l'État. Un certain nombre de chiffres illustrent ce constat. Pour autant, deux bémols sont régulièrement apportés : le vieillissement de la flotte, dont le coût de renouvellement est estimé à 140 millions d'euros, et l'évolution préoccupante de la démographie des bénévoles. Monsieur le secrétaire

Vous avez organisé une table ronde au ministère ; nous y avons participé. Vous avez présenté les résultats d'une enquête menée par les préfets auprès des stations locales SNSM : ceux-ci rejoignent nos conclusions. Enfin, à l'occasion du CIMer, le Premier ministre a évoqué les effets attendus des mesures à engager- voici,

la mesure de l'engagement des bénévoles de cette association. Il a profondément ébranlé toute la communauté maritime. Ce soir, je rends de nouveau hommage aux disparus, à leurs familles, à toutes celles et tous ceux qui agissent pour le sauvetage en mer. mer. Nous leur devons bien plus que des mots : comme l'a dit le Président de la République lors de l'hommage national, « faire vivre ce beau modèle, solidaire et fraternel, du sauvetage en mer », c'est honorer leur mémoire. Et, à ce titre, il faut relever les défis auxquels la SNSM fait face. d'information les souligne parfaitement : pérennité du financement et visibilité face aux besoins de renouvellement de la flotte et de la formation des bénévoles ; pérennisation du bénévolat- les bénévoles veulent aujourd'hui être mieux reconnus, mieux accompagnés et mieux protégés - ; modernisation de la gouvernance de la SNSM, pour préserver le dynamisme de sa structure et sa proximité avec les territoires.

tous ont confirmé leur attachement au modèle original de la SNSM, reposant sur ces trois piliers indissociables que sont le bénévolat, l'autonomie financière et le statut associatif.

C'est d'abord le renforcement du soutien financier de l'État, en portant la subvention annuelle de 6 millions d'euros à près de 11 millions d'euros. C'est aussi l'attribution de la qualité de pupille de la Nation aux enfants

C'est enfin une nouvelle dynamique partenariale entre l'État, la SNSM, les collectivités locales et les bénéficiaires de la SNSM, sur la période allant Ce travail intervient à un moment clé de la vie de l'association, qui connaît une passation de présidence ; je sais qu'il importe à son nouveau président, Emmanuel de Oliveira, de construire, avec tous les membres de la SNSM, une vision stratégique. Ses deux mots d'ordre vont dans ce sens : assurer les capacités opérationnelles et la cohésion. Dans les prochaines semaines, nous devrons stabiliser cette nouvelle dynamique partenariale. Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais partager avec vous quelques-uns des chantiers qui nous attendent.

la trajectoire financière de l'association doit être clarifiée et stabilisée, mais cela passera par l'assurance de l'obtention d'autres ressources financières. Il me vient d'abord à l'esprit l'appui des collectivités territoriales, qui devra se construire en lien avec les associations représentatives, en privilégiant une approche pluriannuelle.

entend amorcer, avec la SNSM, un pacte d'engagement pour les sauveteurs, afin de mobiliser l'ensemble des filières économiques et des usagers bénéficiaires de l'action de l'association. Outre ces deux volets, le paiement des prestations rémunérées assurées par la SNSM doit être facilité. Cela implique un cadre de financement des rapatriements sanitaires consolidé, une meilleure publicité des tarifs des prestations et un recouvrement des paiements

Cet effort sera partagé par les employeurs et les entreprises qui soutiennent l'engagement bénévole. Le Gouvernement sera à leur côté, en proposant un label d'employeur-partenaire de la SNSM et en assurant la promotion des dispositifs existants, comme le congé d'engagement associatif, ou encore le compte d'engagement citoyen. Pour renforcer les équipes techniques, les ministères compétents étudieront aussi les possibilités de recourir à des voies de recrutement alternatives pour certaines fonctions d'appui, comme le service national universel ou le service civique. Enfin, nous accompagnerons l'association dans ses choix de réorganisation.

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Le drame des Sables-d'Olonne, qui a coûté la vie à trois sauveteurs en juin dernier, a rappelé les risques inouïs que ceux-ci prennent pour sauver près de 10 000 personnes par an et en assister bien davantage encore. Dans un département maritime comme le mien, on sait ce que cela signifie.

l'État doit augmenter sa participation, laquelle, je le rappelle, couvre aujourd'hui autour du tiers du budget de la SNSM. Il y va, à notre sens, de la solidarité nationale : l'État ne peut pas être à la traîne du soutien décisif qu'apportent les collectivités locales au fonctionnement de la SNSM. Il importe donc de pérenniser et d'amplifier la rallonge de 4,5 millions d'euros votée dans la loi de finances pour 2020. Plusieurs pistes existent en ce sens, dont un certain nombre ont été rappelées à l'instant par le rapporteur, comme la mise en place d'un prélèvement par les ports de plaisance, la création d'une contribution volontaire à l'achat de navires neufs ou une mise à contribution de la fiscalité sur les permis ou les bateaux de plaisance. Je veux toutefois relever la nécessité de taxer les yachts, mesure qui avait notamment été imaginée pour atténuer l'effet

Vous avez rappelé que le Gouvernement a relevé son soutien annuel de 4,5 millions d'euros, l'établissant à près de 11 millions d'euros, et je porte à votre connaissance que les conditions de trésorerie actuelle de la SNSM sont de nature à satisfaire ses besoins financiers

au travers du pacte d'engagement que j'ai évoqué précédemment pour les sauveteurs et le mécénat, qui pourrait être accru, au regard des pratiques qui ont cours dans certains pays riverains.

En vérité, grâce à la SNSM, cette activité est très peu coûteuse pour l'État. Il apparaît aujourd'hui primordial de préserver la vie des sauveteurs bénévoles tout en consolidant la trajectoire financière de la SNSM pour renouveler une flotte vieillissante. Dans ce processus, il est nécessaire que l'État prenne toute sa part. La mission d'information a relevé l'importance de garantir l'investissement dans les navires, dont la durée de vie avoisine trente ans, par des ressources stables d'État, car le renouvellement de la flotte ne peut rester soumis aux aléas et à la forte variabilité des dons. L'État, en prenant une plus grande part dans l'équipement des stations, leur permettrait de consacrer plus de moyens à l'amélioration de leur fonctionnement et des conditions de vie des bénévoles grâce aux dons qu'elles collectent et aux subventions que les collectivités territoriales souhaitent leur allouer. Monsieur le secrétaire d'État, jusqu'à présent, les ressources perçues par la SNSM lui ont permis, au prix d'une charge excessive pesant sur les stations de sauvetage, de remplir sa mission avec succès et de lancer des programmes de formation des bénévoles et de renouvellement d'une partie de sa flotte d'intervention. La nécessité d'investir fait consensus en raison de l'obsolescence croissante de la flotte actuellement en service et de la nécessité de poursuivre la démarche de qualification des bénévoles.

je rappelle d'abord les obligations issues des traités internationaux qui pèsent sur l'État en matière de veille et à de coordination des secours. J'ajoute qu'à la suite de l'augmentation de la subvention annuelle en 2020 et en incluant les taxes affectées la part de l'État représente aujourd'hui plus de 30 % des ressources de la SNSM, sans compter

secrétaire d'État, mes chers collègues, en cette période d'épiphanie, les habitants de Cherbourg-en-Cotentin, de Landunvez ou de Saint-Malo peuvent soutenir les sauveteurs de la SNSM en achetant des galettes dont les fèves arborent les couleurs des stations de sauvetage. Cette initiative s'ajoute aux nombreuses actions de bienfaisance qui s'avèrent nécessaires pour contribuer au financement d'un service à vocation régalienne. Huit propositions figurent dans le rapport pour garantir sur le long terme le financement des investissements. Pouvons-nous parler de serpent de mer, tant le sujet a été abordé ces dernières années ? Il a été question d'une taxe sur l'éolien en mer, sur le permis côtier, sur l'achat de navires de plaisance

il apparaît clairement que le financement de la SNSM, qui remplit des missions de service public, doit être pris en charge par l'État. Tout en étant consciente de l'effort que le Gouvernement a consenti dans le cadre de la loi de finances, je vous demande, monsieur le secrétaire

hors taxes affectées, qui a vocation à financer en priorité les investissements de la SNSM. Je l'ai dit, un travail va être engagé avec la nouvelle direction de la SNSM pour stabiliser la trajectoire financière et la programmation du renouvellement des moyens ; il pourrait d'ailleurs conduire à revoir la prise en charge des investissements entre le siège de la SNSM, l'État, les collectivités et les stations. L'État est attaché à maintenir une part de financement local dans les projets d'investissement, car cela donne aux stations du poids pour peser dans la décision sur les caractéristiques des moyens nautiques et responsabilise quant à leur format, aux capacités d'armement des navires dans la durée, mais aussi quant à la bonne exploitation du matériel. Le fonctionnement quotidien de la SNSM impliquant un appui des collectivités qui en tirent un bénéfice, il importe donc que celles-ci s'engagent sur les projets d'investissement. Par ailleurs, s'agissant de la sécurité civile, puisque vous y avez fait allusion, je rappelle que l'État finance un certain nombre de matériels, notamment d'hélicoptères et d'avions, qui concourent, d'une manière générale, au sauvetage des personnes. La parole est à M. Jean-François Rapin. Madame Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me permets d'attirer votre attention sur la formation des sauveteurs en mer. Nous comptons de moins en moins d'anciens marins parmi ces sauveteurs bénévoles. Aussi, cette formation permet-elle à ces derniers non seulement d'apprendre la mer, mais également de se familiariser avec les nouveaux bateaux. Lors des Assises de l'économie de la mer qui se sont tenues à Montpellier, le 3 décembre dernier, le Président de la République déclarait souhaiter que le Gouvernement travaille à la reconnaissance, au soutien et à la valorisation des formations qualifiantes dispensées par la SNSM.

que les formations dispensées aux sauveteurs en mer soient éligibles au fonds de la formation professionnelle de France compétences. Le comité interministériel de la mer qui a eu lieu au mois de décembre ne semble pas avoir précisé cette demande de formation cruciale pour le sauvetage en mer. mer. Je salue l'effort budgétaire qui a été réalisé, mais, à mon sens, ces crédits ne suffiront pas à assurer une formation pérenne aux sauveteurs. Par ailleurs, aucun détail n'a été apporté sur l'éligibilité de ces formations à France compétences, alors que, pour la SNSM, cette garantie de financement est indispensable. Qu'en est-il à ce jour ? Enfin, comme je l'ai fait dans le cadre de la mission, j'insiste de nouveau sur le fait que nous disposons, sur les territoires, de lieux de formation de proximité : les lycées maritimes, lesquels dépendent de votre ministère, Les régions en ont la responsabilité et sachez, d'ores et déjà, que la région Hauts-de-France, qui en construira un nouveau prochainement, est disposée à s'engager dans une expérimentation en ce sens.

L'augmentation du soutien financier permettra d'accroître les actions de formation des bénévoles et nous allons accompagner la SNSM, afin de développer, notamment, l'offre de formation de proximité, mais également travailler à la valorisation des compétences et à la reconnaissance des formations dispensées par le pôle national de formation. France compétences sera donc pleinement mobilisée, non seulement pour étudier l'éligibilité de ces formations nécessaires,

dans notre troisième proposition. Il est également nécessaire de clarifier les relations entre le siège et les stations. Notre vingt-deuxième proposition, qui vise à constituer la SNSM en structure fédérale est, de mon point de vue, pertinente. Envisagez-vous de permettre de telles modifications statutaires, monsieur

la prévention ne saurait se limiter à la diffusion des bonnes pratiques, aussi importante soit-elle. L'action de l'État en la matière est primordiale. Entretenir et sécuriser la signalétique de nos littoraux est indispensable à la prévention des accidents maritimes. Dans le Finistère nord, la réforme de la flotte se traduit ainsi par la construction d'un bateau de vingt-huit mètres en remplacement des deux bateaux de dix-sept mètres actuellement en service pour entretenir les phares et les balises du littoral.

Ils s'interrogent également sur la maniabilité d'un tel navire et sur les conséquences que ce changement emportera pour leurs emplois. Il est en outre question de transférer le navire, basé à Morlaix. Si tel devait être le cas, l'entretien des balises du littoral nord-finistérien ne pourrait plus être optimal, puisqu'un navire plus grand ne pourra pas accéder à bon nombre de zones. zones. Je souhaite donc savoir si le Gouvernement entend corriger cette décision, afin de maintenir le parfait entretien des éléments de signalement et de balisage sur la côte et, par conséquent, le niveau de sécurité maritime. La parole maritime. La parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, s'agissant de la signalisation maritime, la réforme que vous évoquez consiste notamment à moderniser la flotte des navires-baliseurs dédiés à l'entretien des ouvrages en mer avec des navires plus performants, plus endurants et permettant d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents tout en optimisant les prestations, les coûts d'entretien et la réduction de la signature environnementale. Certes, nous envisageons bien une réduction du nombre de navires, mais pas au détriment de la qualité du service, puisque ces navires auront un taux d'utilisation plus important et des capacités supérieures de rayon d'action et d'emport. S'agissant de la réforme des services des phares et balises, qui exige, d'ailleurs, un ambitieux plan d'investissement lancé cette année, elle s'inscrit dans une démarche de progrès pour les usagers, avec des ouvrages de signalisation adaptés aux nouveaux besoins des navigateurs, et sera menée

Or la structure de son financement repose à 80 % sur les dons privés, ce qui est incompatible avec la pérennité requise par de tels investissements. Le financement de la SNSM doit donc gagner en visibilité pour garantir que, à l'avenir, ses missions pourront continuer à être assurées efficacement tout en préservant la sécurité des bénévoles et des personnes secourues. S'agissant de la contribution des usagers de la mer, la solution visant à responsabiliser les plaisanciers qui ne disposent pas d'assurance en cas d'intervention, proposée par M. Yves Lyon-Caen, président de la Fédération des industries nautiques, lors de son audition, pourrait constituer une voie intermédiaire intéressante avant la généralisation d'une assurance obligatoire, proposée par la mission d'information. Le recouvrement des créances de la SNSM, lorsque celle-ci intervient en assistance aux biens, doit par par ailleurs être amélioré. Pour ce qui concerne l'assistance aux personnes, si cette mission est exercée par des bénévoles, elle revêt un caractère régalien. La part de l'intervention financière de l'État doit donc évoluer pour couvrir au moins le renouvellement de la flotte de sauvetage en mer et son entretien. le recours à toute création ou réaffectation de taxe doit être pesé. Les activités maritimes ne sont certes pas victimes d'une forte fiscalisation, mais il ne faudrait pas, pour autant, pénaliser les petits plaisanciers. Dès lors, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous préciser l'approche pluriannuelle des engagements de l'État auprès de la SNSM permettant de soutenir les investissements nécessaires ?

telle qu'elle est aujourd'hui envisagée. En revanche, l'assistance aux biens constitue une prestation commerciale qui entre dans le champ concurrentiel. Or l'État ne peut interférer dans des relations commerciales. La SNSM doit donc travailler à une meilleure visibilité des tarifs de ces prestations de remorquage, notamment, et- pourquoi pas

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'an dernier, en France, plus de la moitié des plaisanciers en difficulté, soit environ 20 000 hommes, femmes et enfants, ont été secourus par la Société nationale de sauvetage en mer. Cette contribution considérable à la sécurité maritime est le fait de 8 000 bénévoles qui ont décidé de venir en aide à la vie d'autrui, au risque de perdre la leur. Comme vous le savez, le 7 juin 2019, trois secouristes de la SNSM de la station des Sables-d'Olonne ont péri en mer au cours d'une opération de sauvetage. Ce drame nous a évidemment tous profondément bouleversés. Lors des Assises de l'économie de la mer qui se sont tenues à Montpellier le 3 décembre dernier, le Président de la République leur a rendu hommage avec l'ensemble des acteurs du monde maritime. À cette occasion, il a annoncé que les enfants des secouristes disparus seraient reconnus pupilles de la Nation. La parole de l'État a été partiellement respectée : une semaine plus tard, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la proposition de loi qui accorde la qualité de pupille de la Nation aux enfants de sauveteurs en mer décédés. Nous attendons encore l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Sénat pour marquer définitivement la reconnaissance de la représentation nationale. Grâce à la mobilisation unanime des élus, le Parlement a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, l'augmentation, proposée par le Gouvernement, de 4,5 millions d'euros de la dotation de l'État en faveur de la SNSM, conformément à une demande faite par la mission d'information sénatoriale.

concernant l'attribution rétroactive de la qualité de pupille de la Nation aux enfants de sauveteurs péris en mer lors d'une opération de sauvetage, l'Assemblée nationale a effectivement adopté à l'unanimité une proposition de loi à cet effet le 12 décembre dernier. Le délai constitutionnel d'inscription à l'ordre du jour au

2019, le ministère a versé une subvention de 6 millions d'euros hors taxes affectées à la SNSM et la nouvelle convention pluriannuelle, en cours de rédaction, prévoit un montant alloué de 10,5 millions d'euros au profit de l'association.

revanche, l'État est favorable à la généralisation des assurances pour les navires dans les ports où ils mouillent à l'année, notamment pour prendre en compte le risque lié à l'enlèvement des épaves.

lors, la SNSM des Alpes-Maritimes souhaiterait une plus grande flexibilité lui permettant de proposer elle aussi des formations nautiques dans les lycées maritimes locaux.

la matière, bien au-delà des mots, il faut agir, par exemple en facilitant les heures d'absence des bénévoles auprès de leur entreprise ou de leur administration et en les indemnisant.

obligatoires, si les cotisations sociales devenaient facultatives ? La base de la solidarité, c'est la prise en considération des dangers potentiels que chacune et chacun d'entre nous peut courir.

la reconnaissance de l'engagement et la consolidation de la condition de bénévole seront un aspect fondamental. Comme je l'ai déjà indiqué, nous souhaitons développer l'offre de proximité en matière de formation et nous travaillons déjà à la valorisation des compétences et à la création d'un label « employeur partenaire de la SNSM

au mieux un alignement sur les risques automobiles, c'est-à-dire un contrat d'assurance au tiers, ne couvrant pas le remorquage. C'est pourquoi calquer l'assurance maritime sur l'assurance automobile ne serait pas opérant.

Le dialogue engagé avec le siège de la SNSM a rapidement tourné au monologue. L'un des responsables et son délégué départemental nous ont enjoints à plusieurs reprises de changer nous-mêmes les étiquettes pour indiquer de nouvelles dates de validité, qui permettraient, selon le siège, d'éviter de longues discussions inutiles avec le centre de sécurité des navires. » Incroyable ! Je cite encore Le patron référent de notre station et l'ensemble des bénévoles ont refusé de s'exécuter, préférant privilégier la sécurité par rapport à l'obéissance. » J'en aurais fait autant Ce point d'orgue a conduit le président de notre station, son vice-président, son patron référent, un patron suppléant et quatre canotiers, soit un tiers de la station, à démissionner durant la première quinzaine du mois de décembre 2019. Le sous-préfet de Saint-Paul est informé et très surpris.

peine à trouver des financements pour le renouvellement des canots de sauvetage et l'entretien des matériels. Une des propositions du rapport de Didier Mandelli consiste à faire évoluer la gouvernance de la SNSM. De fait, une association de la société civile composée de bénévoles engagés et dévoués,

principe démocratique fondamental, le président et les principaux dirigeants élus de la SNSM doivent l'être en toute transparence et d'une manière démocratique. C'est devenu une exigence,

d'État, vous interroger sur la sécurisation des financements de la SNSM, enjeu d'une particulière acuité. Comme il a été souligné à plusieurs reprises, la SNSM, l'une des institutions les plus respectées du monde associatif, remplit une véritable mission de service public, grâce à ses 8 000 sauveteurs bénévoles répartis sur plus de 200 stations, qui interviennent nuit et jour, été comme hiver, pour porter secours aux personnes en péril en mer. En 2018, plus de 10 000 personnes ont ainsi été secourues par les sauveteurs en mer, et plus de 20 000 ont bénéficié de leurs soins. Pourtant, alors que la survie de ce modèle nous concerne tous, la SNSM ne dispose toujours pas des moyens suffisants pour lui permettre d'assurer le nécessaire renouvellement de sa flotte de sauvetage et la formation de ses sauveteurs. Ainsi appelle-t-elle régulièrement à la mobilisation de l'État, des collectivités territoriales mécènes et des donateurs individuels. En ce qui concerne l'engagement financier de l'État, au-delà des discussions budgétaires de la fin de l'année dernière,

Depuis lors, le trafic maritime s'est développé avec des gros porteurs, mais aussi autour du loisir et des sports nautiques, ce qui a modifié sensiblement

des baignades. La SNSM exerce d'autres missions, qui sont des activités rémunérées et qui relèvent de la sphère commerciale et concurrentielle : l'assistance et le remorquage en mer, la surveillance des manifestations, la dispersion des cendres en mer. L'État, par sa subvention annuelle, soutient la SNSM dans sa mission de sauvetage en mer. Le modèle particulier du sauvetage en mer a été confirmé. Il repose sur les piliers- je les ai rappelés il y a un instant -que sont le bénévolat, le statut associatif et l'autonomie financière résultant

À vous entendre, j'ai vraiment l'impression que vous vous satisfaites de la situation présente. J'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas lu le rapport de M. Mandelli. Et j'ai vraiment l'impression que, dans un an, en espérant que, d'ici là, il n'y aura pas

En 2017, l'État attribuait le label « grande cause nationale » à la SNSM, reconnaissant ainsi unanimement l'engagement et l'abnégation des 8 000 sauveteurs bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour sauver les usagers de la mer en détresse. Cette mission de service public exigeante impose à ces bénévoles de nombreux sacrifices pour parvenir à concilier leur vie professionnelle, personnelle et associative. Que ce soit pour la surveillance des plages ou pour le sauvetage en mer, les missions exercées par les sauveteurs bénévoles sont de plus en plus nombreuses, longues et techniques. Elles mobilisent des compétences diverses et imposent un niveau de formation en constante augmentation pour garantir le niveau de performance exceptionnel qu'est celui de la SNSM, d'autant que de moins en moins de bénévoles sont directement issus du monde maritime. Aujourd'hui, les formations sont réalisées soit directement dans les stations, dans les trente-deux centres de formation et d'intervention comme celui du Havre, soit, pour les formations les plus qualifiantes, au pôle de formation de Saint-Nazaire, sans oublier

la gratuité reste souvent théorique. Comment assurer la prise en compte de la validation des acquis de l'expérience, notamment pour ceux qui sont formés sur le tas, la transmission du savoir-faire

Afin de mieux l'organiser, l'État a validé un nouveau diplôme de sauveteur secouriste aquatique en milieu naturel. Sa généralisation a cependant été différée face aux difficultés des communes, confrontées à la pénurie du recrutement. De plus, le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA), dont les sessions d'examen étaient jusqu'alors organisées par les services de l'État, est depuis le 1janvier sous la responsabilité des associations agréées agréées de sécurité civile, qui sont elles-mêmes déjà chargées de la formation des candidats. Si ces réformes vont dans le sens de la responsabilisation et de la valorisation des bénévoles des associations, celles-ci hésitent à s'engager dans ces nouveaux processus de formation et d'habilitation, parce qu'elles ne comprennent pas l'articulation entre le BNSSA et le diplôme de sauveteur secouriste aquatique en milieu naturel. Monsieur le secrétaire d'État, ne serait-il pas nécessaire d'accélérer la réforme du BNSSA, dont le contenu est peu adapté aux besoins réels de formation des sauveteurs côtiers, et d'en faire un diplôme de sauveteur secouriste aquatique en milieu artificiel, de préciser le rôle du diplôme de sauveteur secouriste aquatique en milieu naturel en l'inscrivant dans le code général des collectivités locales et le code du sport ? Bref, n'est-il pas urgent de clarifier l'adéquation entre diplômes et compétences requises en fonction des milieux d'exercice ? ? La parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous avez rappelé que, durant la saison estivale, les nageurs sauveteurs employés et rémunérés par les communes sont déployés dans plus de 260 postes de secours, ce qui permet d'assurer la surveillance de plus d'un tiers des plages métropolitaines. La participation à cette mission de surveillance et de sauvetage implique, pour les nageurs sauveteurs, de suivre une formation de haut niveau, dispensée dans les trente-deux centres de formation et d'intervention de la SNSM, qui couvrent l'ensemble du territoire et fonctionnent grâce à l'implication des instructeurs bénévoles. Ces derniers consacrent chaque année plusieurs dizaines de journées d'engagement bénévole au service de la qualification des jeunes nageurs sauveteurs. Les stages de formation suivent des référentiels qui sont définis à la fois par l'État pour la formation aux premiers secours, le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, le BNSSA, et le permis côtier, et le permis côtier, et par la SNSM. Même si des évolutions peuvent être envisagées, je crois que, aujourd'hui, ils sont cohérents les uns par rapport aux autres. Et fort de cette formation de qualité, les nageurs sauveteurs de la SNSM forment un vivier de recrutement de choix pour les maires des communes littorales. Ils sont progressivement devenus des acteurs incontournables pour l'exercice des missions de surveillance et de sauvetage des plages.

Nous avons abordé un sujet qui nous tient tous à coeur et qui réunit, d'une part, des préoccupations liées à la sécurité des usagers de la mer, aux moyens que nous y consacrons et, d'autre part, des enjeux humains qui touchent à l'engagement total et gratuit de femmes et d'hommes qui méritent notre admiration et notre soutien. Je veux ici leur rendre hommage. Je tiens aussi à exprimer l'honneur et le réel plaisir que j'ai eus à présider cette mission commune d'information aux côtés du rapporteur Didier Mandelli, et de tous les collègues membres de la mission, qui ont été particulièrement présents et ont largement participé à l'organisation de nos déplacements sur le littoral métropolitain et ultramarin. Comme ce fut le cas dans mon département, le Calvados, où nous nous sommes rendus à la fin du mois d'août, je sais que les sauveteurs que nous avons rencontrés dans les stations et les centres de formation les centres de formation ont été très sensibles au fait que nous venions les entendre sur les lieux mêmes où ils exercent leur mission. Je pense que nous avons rempli notre mission. libéré la parole des bénévoles que nous sommes allés voir prioritairement, avant de recevoir les acteurs institutionnels. Nous avons également abordé publiquement certains sujets relatifs au fonctionnement, aux circuits administratifs et financiers de la SNSM, qui n'étaient pas réellement traités dans les précédents rapports administratifs. En exposant certains travers du système actuel, souvent méconnus de nos concitoyens, comme le poids excessif qui pèse sur les bénévoles des stations pour le financement de leur matériel, nous n'avons pas menacé l'organisation du sauvetage en mer. Bien au contraire, nous pensons aider à sa pérennisation sur des bases plus saines et adaptées à notre temps. Aussi, et c'est à souligner, notre mission commune d'information a travaillé rapidement et rendu ses conclusions trois mois et demi après sa constitution. Nous voulions être en mesure de présenter notre constat et nos propositions avant le rendez-vous annuel qui détermine la politique nationale dans le domaine maritime, et de contribuer ainsi à la définition des orientations. Nous aurions aimé échanger avec le Gouvernement avant la remise du rapport, mais notre invitation à entendre la ministre chargée du dossier ne s'est pas concrétisée, n'ayant pas été acceptée. Le comité interministériel de la mer (CIMer) s'est réuni le 19 décembre dernier, quelques jours après le discours du Président de la République aux assises de l'économie de la mer de Montpellier. le Gouvernement a dressé un constat que nous partageons : les bénévoles souhaitent être mieux reconnus, mieux accompagnés et mieux protégés. La trajectoire financière doit être stabilisée et la gouvernance rénovée. Trois mesures ont été actées dans ce cadre. La première consiste à accompagner la pérennisation du modèle économique de l'association en portant à 10,5 millions d'euros le soutien financier de l'État.

La deuxième mesure est l'attribution de la qualité de pupille de la Nation aux enfants de sauveteurs en mer péris lors d'opérations de sauvetage, avec effet rétroactif. Cette disposition a fait l'objet d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 12 décembre dernier et transmise le même jour à notre assemblée. s'agit effectivement d'une bonne mesure, mais elle est loin de satisfaire toutes les justes demandes des bénévoles. Elle ne saurait bien entendu à elle seule résumer ce qui est attendu au titre de l'amélioration et de la clarification de la condition de bénévole. La troisième mesure nous intéresse encore plus, car elle se rapproche de notre préoccupation centrale dans ce dossier, à savoir la gouvernance de la SNSM. Il s'agit de définir et d'entériner un plan d'action partenarial entre l'État, la SNSM et d'autres acteurs, tels que les collectivités locales ou les financeurs à l'horizon de 2020. Le rapporteur a présenté les nombreuses propositions de la mission sur ce sujet. Elles concernent l'organisation interne de la SNSM, qui est bien sûr une association, mais qui pourrait entendre les messages réformateurs que lui adresserait le Gouvernement. Elles concernent plus largement tout l'environnement institutionnel et social autour du sauvetage en mer : les relations avec les collectivités, la sensibilisation des usagers de la mer, et pas seulement des plaisanciers.

d'État, vous comprendrez que nous sommes restés sur notre faim avec le CIMer 2019 et que nous attendons les mesures concrètes que vous pourrez mettre en oeuvre dans le cadre d'une contractualisation avec la SNSM. Même si la mission commune d'information a rendu son rapport, nous ne considérons pas, du côté du Sénat, que le sujet soit clos. Nous sommes tout à fait disposés, si vous le souhaitez, à participer à la définition de nouvelles règles de fonctionnement sur la base de davantage de décentralisation et de démocratie dans les procédures de décision.